Monsieur le président,

La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

et nourris. Je veux remercier mon homologue Laurent Saint-Martin, rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, de son écoute- nous travaillons dans des conditions difficiles, et vous imaginez quels échanges il faut pour arriver à un texte commun.

Certains avaient été votés ici même par de larges majorités ; d'autres sont issus du texte de compromis que nous avons souhaité ensemble, députés et sénateurs, adopter.

d'exonération de l'impôt sur le revenu applicable aux rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires. Pendant cette crise, personne n'en disconviendra, de nombreux salariés

du forfait au-dessous duquel les heures supplémentaires ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Ce plafond est augmenté de moitié pour être porté à 7 500 euros.

en ouvrant les débats, l'image de la bouée de sauvetage qu'il fallait donner à nos entreprises et à nos entrepreneurs. Pour renforcer le plan de soutien aux entreprises, nous avons introduit,

ou de monter au capital de telle ou telle entreprise pour la sauver, il est important qu'un contrôle du Parlement soit prévu. C'est le dispositif du Sénat qui a été retenu, je le répète,une information préalable

des résultats pour le moins singuliers. L'assurance est normalement la garantie d'un aléa, et l'aléa disparaît si l'on ne peut plus circuler ... Nous avons en quelque sorte décidé de faire confiance aux négociations qui s'engagent entre le Gouvernement et les assureurs.

sans doute au cours du mois de mai, en tout cas très prochainement, pour un PLFR n° 3. J'espère qu'il sera consacré à la relance post-déconfinement, mais nous serons sans doute, malheureusement, dans l'obligation de réviser un certain nombre de chiffres- je pense en particulier

d'abord, le financement du chômage partiel passe de 8 milliards d'euros à près de 27 milliards d'euros, financés aux deux tiers par le budget de l'État et à un tiers par l'Unédic, pour préserver la situation des salariés. De ce fait, le relèvement du plafond d'emprunt de l'Unédic garanti par l'État passera de 7 à 10 milliards d'euros.

Si nous devions manquer de crédits pour financer les aides aux entreprises, nous disposerions, entre autres, des crédits mis en réserve sans être affectés, à hauteur de 1,7 milliard d'euros. Par ailleurs nous reviendrions vers vous avec un troisième texte financier.

de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous avons abondé le fonds de développement économique et social (FDES). Rechargé pour atteindre 1 milliard d'euros, il sera mobilisé pour accompagner les entreprises.

À ce jour, le montant des reports d'échéances fiscales s'élève à plus de 4 milliards d'euros et à plus de 12 milliards d'euros pour les échéances sociales. Ce sont donc 16 milliards d'euros qui permettront d'alléger la trésorerie des entreprises concernées. Nous remboursons, en outre, de manière accélérée les créances des entreprises restituables en 2020

et la fin de l'état d'urgence sanitaire, dans un plafond de 7 500 euros, comme l'a souligné le rapporteur. Les secteurs fragiles seront accompagnés plus fortement : 19 millions d'euros sont accordés aux parcs zoologiques, aux refuges et aux cirques familiaux au titre des soins prodigués aux animaux. Ce dispositif sera complété pour apporter un soutien aux centres équestres accueillant du public. Les bailleurs dont les locataires sont des professionnels, que nous avons invités à ne pas percevoir les loyers qui leur reviennent, pourront déduire de leurs revenus imposables les sommes auxquelles ils ont renoncé. C'est une initiative de l'Assemblée nationale, que nous avons soutenue.

utile. La production et l'acquisition des matériels de protection sanitaire ont été facilitées. D'une part, des mesures budgétaires ont été prises pour soutenir l'investissement dans les machines permettant la production de matériaux utilisés pour la confection des masques et d'autres équipements.

subventions. Pour soutenir la solidarité, le plafond des dons alimentaires et de première nécessité donnant droit à un avantage fiscal passera d'un peu plus de 500 euros à 1 000 euros. Je tiens à remercier l'ensemble des parlementaires,

à l'égard de tous, et non pas uniquement d'un programme de sauvetage de notre économie, même si ce dernier point est important. Je me félicite aussi des apports du Sénat, qui sont significatifs.

besoins de nos entreprises pour passer ce cap difficile. Je constate que le Gouvernement a parfaitement écouté les remontées du terrain, provenant à la fois des parlementaires, des organisations professionnelles et des entreprises,

Nos débats n'ont pas bouleversé cette stratégie. Les amendements n'ont ni supprimé ni remplacé des mesures adoptées : ils les ont complétées, améliorées,

a apporté plusieurs modifications intéressantes : il a notamment complété le dispositif voulu par l'Assemblée nationale d'une TVA réduite à 5,5 % pour certains types de produits en y ajoutant les équipements de protection sanitaire, élargi les missions du comité de suivi en y intégrant le fonds de soutien

Cette relance devra nécessairement être européenne, parce que nous avons besoin de la solidarité européenne. Elle devra aussi être écologique- à cet égard,

me paraît aller dans le bon sens. Nous avons encore le temps pour le faire ensemble et j'espère que nous le ferons dans le même esprit. Comme le notait Paul Valéry dans ses : « Il faut juger à froid et agir à chaud. » Nous sommes encore dans le temps de l'action à chaud ; très vite viendront le jugement et la réflexion qui pourra permettre à chacun de contribuer et de densifier la relance à venir. Comme l'ordre de marche proposé par le Gouvernement

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, la commission mixte paritaire s'est accordée voilà quelques heures sur un projet de loi de finances rectificative que nous n'approuverons pas. Au cours des débats de ces derniers jours, nous avons relevé les manques criants de ce texte et formulé de nombreuses propositions. À chacune d'entre elles, ou presque, le Gouvernement et la commission des finances nous ont répondu : ce texte est un texte d'urgence, nous renvoyons le débat de fond à plus tard. En quelque sorte, l'heure serait non pas au débat politique, mais à l'action. Nous réfutons totalement ce point de vue

Or l'après se pense, se débat, se prépare, s'organise pendant. Pourquoi vouloir mettre le couvercle sur le débat contradictoire au nom de l'urgence ? pas question de contester les options profondément libérales que vous maintenez au nom de cette urgence ? Un autre argument est invoqué pour voter ce texte, celui de la responsabilité. Cet argument est pour nous totalement irrecevable. Ainsi, même en doutant de la démarche gouvernementale face au rejet de l'essentiel de nos propositions, il faudrait voter pour, « en responsabilité

une mise au pas. Nous avons un avis différent. Nous l'assumons ici, mais aussi devant le peuple. J'insiste sur ce dernier point : nous ne sommes pas dans une bulle ; les citoyens écoutent ce qui est dit ils réfléchissent ; même confinés, ils expriment des opinions. Un sondage publié mardi dernier était d'ailleurs édifiant quant à la défiance à l'égard de l'action gouvernementale. L'Assemblée nationale et le Sénat débattent, et c'est une bonne chose. Il faut avoir le courage de s'opposer, lorsque l'on estime que les valeurs que l'on défend sont remises en cause. L'opinion évolue, est attentive ; la situation évolue aussi.

Vous avez rejeté, comme aux plus beaux jours de la présidence des riches, toutes nos propositions d'une participation accrue des plus fortunés de la solidarité nationale. Rétablir l'ISF ? C'est toujours non ! Supprimer le prélèvement forfaitaire unique ? Non ! Augmenter la contribution des plus hauts revenus ? C'est encore non

Pouvez-vous nous indiquer si l'État prend en charge ce chômage partiel ? Être responsable, c'est déterminer qui va payer la dette, ce qu'elle va devenir. Allez-vous continuer à casser le service public, à contraindre les plus défavorisés ? Votre rejet de nos propositions de justice fiscale le laisse craindre. Le débat parlementaire est incomplet. Vous annoncez 20 milliards d'euros de participation financière de l'État pour aider les entreprises stratégiques en difficulté.

donc pas question pour nous de valider ainsi une opération de secours aux actionnaires défaillants pour leur rendre la maison assainie dès la crise passée. Nos amendements visant à améliorer le sort des plus démunis,

Un mois après la première loi de finances rectificative, le Parlement autorise de nouveau le Gouvernement à déployer des moyens massifs et sans précédent pour venir en aide à toutes les entreprises et à tous les secteurs en difficulté. Nous partageons pleinement la logique de ce deuxième volet du plan d'urgence pour soutenir et rendre possible la reprise de notre économie. Je me réjouis que nous ayons pu trouver un terrain d'entente avec nos collègues députés : cela permettra une mise en application rapide de ces nouveaux dispositifs. L'investissement collectif est massif et même sans précédent, mais la dépense publique atteint de nouveaux records, tant en valeur absolue qu'en proportion de la richesse nationale, alors que, dans le même temps, la recette publique chute brutalement, le déficit se creuse et la dette explose. Aussi, je tiens à rappeler à cet instant que nous finançons aujourd'hui un plan de sauvegarde nécessaire de notre économie avec de l'argent que nous n'avons pas. Cet effort reposera sur les générations futures. Pour rétablir nos finances publiques, nous aurons besoin de toutes nos entreprises et d'une France mobilisée et rassemblée. Nous aurons besoin de nos grands groupes, dont certains seront recapitalisés par l'État, si c'est nécessaire, et qui devront se transformer. Nous aurons besoin de nos ETI, qui recourent largement au chômage partiel, de nos PME, qui qui ont pu bénéficier de prêts garantis par l'État, de nos artisans et indépendants, qui seront soutenus par le fonds de solidarité, de nos agriculteurs, confrontés à la crise- certaines filières, comme celles des biocarburants ou de l'horticulture, nécessiteront des mesures supplémentaires. Je salue également l'activation hier par la Commission européenne des mécanismes de crise, tels que la gestion des stocks privés et la flexibilité financière. Les mesures adoptées voilà un un mois ont commencé à faire leurs preuves. Aujourd'hui, nous les améliorons et nous les renforçons. Notre priorité doit rester la santé des Français et la préservation du tissu économique et social. notre modèle social est mis à rude épreuve par cette crise. C'est pourquoi nous devons dès maintenant nous focaliser sur la reprise économique et trouver les moyens de la financer à long terme en mobilisant toutes nos forces. Je relève des points de satisfaction importants retenus sur proposition du Sénat. Je pense à l'augmentation de la défiscalisation des heures supplémentaires, au renforcement des dispositions, dites loi Coluche, pour soutenir la générosité des Français, mais également aux 8 millions d'euros supplémentaires en direction des 3 400 communes de moins de 500 habitants, qui sont particulièrement engagées dans cette crise. revanche, l'annulation des charges et cotisations sociales pour les entreprises les plus en difficulté reste en suspens et devra faire l'objet de discussions à venir. Il en va de même de la contribution des assureurs et de la non-éligibilité au dispositif de solidarité nationale des entreprises liées à des paradis fiscaux, comme nous l'avions proposé. Le déconfinement apparaît aujourd'hui comme un enjeu essentiel : il faudra faire preuve de méthode et aussi s'appuyer sur les élus locaux. nous nous mobilisons désormais au Sénat pour être au rendez-vous de ce plan de relance. Celui-ci devra s'appuyer là aussi sur les collectivités territoriales, qui font preuve d'une mobilisation et d'une efficacité exceptionnelles du fait de leur proximité territoriale. de cette crise que la France a besoin d'un État plus décentralisé, qui puisse agir au plus près des territoires, bref, d'une vision renouvelée des libertés locales et de la décentralisation. Nous voterons bien évidemment les conclusions de la commission

la commission mixte paritaire qui s'est tenue à midi sur ce deuxième projet de loi de finances rectificative a abouti à un accord. La chose est suffisamment rare en matière de loi de finances pour que nous nous en réjouissions. Cet accord est une bonne nouvelle pour le pays après débat, bien sûr avec des nuances, la représentation nationale sait nouer les compromis nécessaires pour faire face à l'urgence sanitaire et économique, et de premières dispositions sociales sont prises. Le contexte est exceptionnel : les inconnues sont nombreuses et les données économiques chaque jour fluctuantes. Nous savons ce texte attendu par tous ceux que la pandémie de Covid-19 expose aux pires difficultés. Dans un esprit de responsabilité, députés et sénateurs ont su travailler en bonne intelligence, avec pour seul souci la préservation du tissu productif français et la reconnaissance de ceux qui, parfois au péril de leur vie, affrontent avec courage le danger du coronavirus. Il fallait faire la part entre l'urgence- le soutien aux soignants, à l'emploi et au tissu économique -, la nécessaire attention à des secteurs d'activité dont la situation nous semblait insuffisamment prise en compte et la conscience que tout cela doit « se phaser » dans le temps et qu'il y aura bien sûr un PLFR 3

Encore ces chiffres restent-ils suspendus à une aggravation que d'aucuns nous prédisent. Il y aura un débat sur la façon de rembourser cette dette, qui se creuse dans des proportions abyssales, et de réduire l'impact du choc sur nos comptes publics. Les motifs de satisfaction du groupe Union Centriste sont nombreux. La commission mixte paritaire a ce matin commencé sous les meilleurs auspices, après que Bruno Le Maire a annoncé l'exclusion des aides publiques pour les entreprises ayant leur siège dans un paradis fiscal. Cela Cela faisait suite à l'adoption par la Haute Assemblée de notre amendement, déposé sur l'initiative de notre collègue Nathalie Goulet. C'est là une clarification bienvenue : aucune entreprise violant le pacte social ne doit profiter de la solidarité nationale. Dommage que cette disposition ne figure pas dans les

devant les maires des petites communes, qui font aujourd'hui preuve d'un engagement et d'une détermination sans faille. Cette avancée a pu être obtenue grâce au travail de notre collègue Sylvie Vermeillet, que je tiens à féliciter au nom de l'ensemble de mes collègues centristes. Je m'associe à elle pour saluer l'écoute et le travail fructueux des deux rapporteurs généraux, Albéric de Montgolfier et Laurent Saint-Martin. De la même façon, nous nous félicitons de l'élargissement du taux réduit de TVA à l'ensemble des équipements de protection.

et sociale des heures supplémentaires. Beaucoup de nos compatriotes travaillent durement, et plus durement encore durant la crise sanitaire, le plus souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Ce surcroît Ce surcroît d'effort devait être récompensé. Il le sera grâce à l'accord obtenu en commission mixte paritaire. Nous avons par ailleurs entendu l'explication du Gouvernement concernant la contribution des assurances à l'effort de redressement. Nous espérons que les discussions en cours aboutiront à une solution. Bien sûr, des motifs de regrets demeurent et la perspective déjà proche d'un troisième PLFR sera peut-être pour nous l'occasion de remettre l'ouvrage sur le métier. Je songe aux aux amendements de notre collègue Annick Billon, concernant la création de fonds d'urgence de lutte contre les violences intrafamiliales et d'aide à la parentalité. L'urgence de la crise économique ne doit pas nous faire perdre de vue les urgences non moins imminentes sur le front social. d'autres propositions défendues par nos collègues continueront de retenir notre attention dans les semaines qui viennent. C'est le cas de la question du remboursement du FCTVA ou de celle des délais d'engagement et de clôture des opérations locales d'investissement, posées par nos collègues Michel Canevet et Bernard Delcros. C'est le cas encore de l'imputation en section d'investissement des contributions de l'ensemble des collectivités au fonds national de solidarité, soulignée par Hervé Maurey. Gageons aussi que, d'ici au prochain collectif budgétaire, la transformation du report des échéances sociales et fiscales en annulation pour les entreprises les plus affectées deviendra une réalité. Des négociations sont en cours et nous souhaitons que le Gouvernement parvienne à soulager les entreprises gravement affectées par la crise. Plusieurs amendements préfiguraient un plan de relance d'urgence et ont été écartés à ce titre. Nous disons au Gouvernement qu'il nous faudra construire collectivement ce plan de relance et d'investissement. Dans l'immédiat, nous saluons la diversité et la montée en puissance des dispositifs présentés voilà un peu plus d'un mois par le Gouvernement et nous adopterons à l'unanimité ce deuxième projet de budget rectificatif enrichi par le Parlement. Je salue chacun de ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce texte, en particulier les membres de la commission des finances, mais aussi l'ensemble des services du Sénat, dans ce contexte si particulier et dans le respect des règles sanitaires. La parole

loi de finances rectificative qui nous a été présenté. La confiance ne se décrète pas. La peur n'est jamais bonne conseillère. Nos chercheurs, nos personnels de santé, nous industriels, nos salariés du front à qui tous les soirs nos concitoyens disent merci donnent de l'espoir. Nous ne devons pas les décevoir. Les amendements défendus par mon groupe avaient pour objet d'ouvrir des débats sur les nécessaires mesures de solidarité à adopter, tout en ne faisant pas reposer leur financement sur la seule dette. Certains de nos concitoyens aux capacités contributives importantes ont bénéficié d'avantages fiscaux importants ; nous considérons qu'ils peuvent participer à l'effort national. Ce fut le sens des propositions concernant l'ISF 2.0, cher au président de la commission des finances, ou le retour à une taxation du capital. Toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Il en va ainsi de notre approche sur le secteur des assurances. amendements que nous avons soutenus ont permis soit d'ouvrir des débats, en proposant des fonds de soutien à des secteurs particulièrement affectés- tourisme, restauration, culture, événementiel, Français de l'étranger soit de conforter les annonces de membres du Gouvernement, en créant des fonds d'urgence pour lutter contre les violences intrafamiliales et aider à la parentalité ou en prévoyant le versement d'une prime exceptionnelle pour les assistants familiaux de l'aide à l'enfance, soit d'aborder la Il faut saluer certaines avancées pour les collectivités territoriales, qui doivent gérer le quotidien. Ainsi, la baisse du taux de TVA à 5,5 %, élargie à tous les produits de protection contre le Covid-19, est une bonne chose. Nous ressentons toutefois à l'abandon d'amendements que nous considérions comme un premier pas pour rétablir une certaine solidarité. Monsieur le rapporteur général, j'ai pris acte de votre vigilance concernant le secteur des assurances. Mon groupe ne renoncera pas à son ADN de justice sociale et fiscale. Les prochains plans de sortie du confinement et de relance, qui ne manqueront pas d'advenir, nous trouveront vigilants et combatifs sur ce point et sûrement moins conciliants. de même en ce qui concerne les annonces de ministres non suivies d'effet ou les amendements, notamment du rapporteur général, visant à abonder de 2 milliards d'euros le fonds de solidarité pour les entreprises, à la suite de la crise sanitaire.

afin de soutenir le chômage partiel, qui touche plus de 10 millions de nos concitoyens, et nos entreprises. N'ajoutons pas à la crise sanitaire une crise économique que nous ne souhaitons pas voir se transformer en crise sociale, nos concitoyens les plus modestes étant déjà profondément affectés, ne serait-ce que pour se nourrir. Chaque jour qui passe conduit inexorablement au monde d'après

pour lesquelles nous demandons l'annulation des charges sociales et fiscales parce qu'elles ne pourront pas reprendre leurs activités le 11 mai ou parce qu'elles ont perdu du jour au lendemain,

qui engagera le débat pour tenter d'apporter des solutions. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas rester les bras ballants. Nous regrettons aussi, monsieur le secrétaire

payée par les collectivités locales sur les achats d'équipements de protection individuelle le fonds de compensation de la TVA. Les collectivités locales ont simplement cherché à pallier les carences de l'État en matière d'importation de masques.

loi de finances rectificative. Je pense à la hausse du plafond concernant les heures supplémentaires pour les salariés et les fonctionnaires qui sont en première, deuxième ou troisième ligne sur le terrain. pense ensuite au prêt participatif adossé au FDES pour les très petites entreprises et les PME, qui parfois se voient refuser par leur banque un prêt garanti par l'État. Je pense aussi à l'encouragement fiscal au don vis-à-vis des

du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.